La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 4 avril 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté.

la Réunion. Ce projet d'outil multifilières de traitement des déchets, qui développe la valorisation matière puis énergétique des déchets, est responsable puisqu'il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre produit par les déchets. Il intègre pleinement les objectifs de la feuille de route nationale de l'économie circulaire et la stratégie nationale bas-carbone en cours de révision, avec laquelle doivent être compatibles les programmations pluriannuelles de l'énergie, ou Il est entièrement conforme aux orientations nationales et européennes en matière de stratégie pour l'énergie et le climat, en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre et à la décarbonation de l'énergie promue

du territoire réunionnais, en réduisant la pollution des sols, de la mer, des rivières, en luttant contre la prolifération des maladies à transmission vectorielle et en réduisant les émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre.

Toutefois, comme vous le savez, madame la secrétaire d'État, la PPE de La Réunion est actuellement en cours de révision et le porteur du projet ne dispose pas d'informations sur l'avancée et le contenu de cette révision. Or cette situation est susceptible de paralyser le projet d'Ileva. En effet, la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, saisie en octobre 2018 du projet de contrat d'achat relatif à l'électricité produite par la valorisation des déchets issus de l'outil multifilières, semble refuser de se prononcer avant de savoir si le projet sera maintenu dans la nouvelle PPE de La Réunion. Je souhaiterais donc vous entendre me confirmer que le maintien de la valorisation énergétique des déchets reste un objectif de développement des énergies renouvelables dans les PPE pour la période 2023-2028.

que le prévoit le code de l'énergie, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, de La Réunion doit être révisée. Cette révision s'inscrit dans un cadre spécifique aux territoires ultramarins. En effet, en premier lieu, chaque territoire dispose d'une programmation pluriannuelle de l'énergie spécifique.

ou les enjeux particuliers autour de la mobilité, qui représente 70 % de l'énergie finale consommée à La Réunion. Sur ces sujets, les importants travaux menés depuis septembre 2017 entre l'État et la région ont permis d'avancer vers une réelle décarbonation du mix énergétique, notamment avec la conversion des centrales à charbon à la biomasse et un ambitieux plan de développement du photovoltaïque. Dans le cadre de cette révision, vous m'interrogez sur le volet relatif au développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables issues de la filière déchets.

La gestion des déchets sur l'île est organisée autour de deux bassins de vie. Pour le moment, chaque bassin prévoit d'implanter sur son territoire une installation de valorisation énergétique à partir de combustibles solides de récupération.

à court et moyen terme. Sans remettre en cause l'objectif de la région, je souhaite qu'une réponse puisse être apportée, sans attendre 2030, à la problématique des déchets à La Réunion. La PPE révisée devra intégrer cette orientation de l'État.

secrétaire d'État, je souhaiterais attirer votre attention sur le refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont ont fait l'objet, ces dernières années, les communes du département d'Indre-et-Loire, fortement touché par les risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Chaque année, des milliers de propriétaires constatent l'affaissement et la déstructuration progressive des murs qui se fissurent gravement, rendant impossible Or, depuis 2011, aucune commune d'Indre-et-Loire n'a été reconnue en état de catastrophe naturelle, sauf un infime pourcentage en 2017. Les refus répétés de l'État ont conduit 35 communes de mon département à se regrouper au sein d'une association, l'association des communes en zone argileuse.

Elle analyse l'intensité des mouvements de terrain différentiels au regard de deux critères : un critère géotechnique, la nature du sol d'assises des constructions doit être sensible au phénomène de retrait-gonflement ; et un critère climatologique, les niveaux d'humidité des sols superficiels doivent faire état d'une sécheresse des sols particulièrement marquée. La méthode scientifique de mise en oeuvre et d'évaluation de ces deux critères, qui n'a aucune existence légale, reste inconnue. En mars 2018, Mme la ministre Gourault a indiqué à notre collègue Nicole Bonnefoy que le caractère normal ou non de l'intensité de l'épisode de sécheresse était apprécié au regard des épisodes de sécheresse ayant précédemment touché le même département. Aussi, alors que le caractère argileux d'un territoire est parfaitement connu et reconnu, la multiplication d'épisodes de sécheresse a nécessairement pour conséquence de normaliser le phénomène. Cette situation est injuste. Mme Gourault a précisé que des réflexions étaient en cours pour définir réglementairement les modalités d'instruction des dossiers de reconnaissance en catastrophe naturelle. En l'absence d'avancée, le Sénat a, il y a quelques semaines, constitué une mission d'information pour identifier les difficultés liées à l'indemnisation des sinistres résultant des aléas naturels de forte intensité et proposer des solutions. Aussi, je souhaiterais savoir où en sont les réflexions pour définir un cadre réglementaire précis et pertinent permettant aux sinistrés d'être indemnisés. J'invite également le Gouvernement à examiner chacune des demandes des communes d'Indre-et-Loire et à leur accorder le bénéfice de l'état de catastrophe naturelle au titre de 2018. La

un épisode de sécheresse des sols a touché le territoire métropolitain au cours du second semestre 2018, notamment dans le nord-est du pays. Au 1 avril 2019, plus de 3 500 demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2018 ont été déposées.

Ensuite, compte tenu de la cinétique lente qui caractérise l'aléa sécheresse et des connaissances scientifiques disponibles à ce jour, deux critères cumulatifs sont mis en oeuvre pour caractériser son intensité une condition géotechnique, un sol d'assise des constructions constitué d'argile sensible aux phénomènes de retrait et/ou de gonflement ; deuxièmement, une condition de nature météorologique, une sécheresse du sol d'intensité anormale. Ce modèle permet à l'autorité administrative d'instruire l'ensemble des demandes sur le fondement de données techniques présentant les mêmes qualités et, ainsi, de s'assurer d'une égalité de traitement des dossiers. L'instruction effective des dossiers déposés au titre de l'année 2018 interviendra au cours du printemps 2019, Météo-France et les services de l'État concernés ayant été sensibilisés à la nécessité de traiter ces demandes dans des délais S'agissant de la simplification de la procédure, elle aboutira dans les prochaines semaines. Les nouveaux critères seront d'ailleurs utilisés dès cette année pour analyser les demandes au titre de l'épisode de sécheresse des sols de l'année 2018. Ces travaux visent deux objectifs : d'abord, prendre en compte l'amélioration des connaissances scientifiques relatives au phénomène, notamment les modalités techniques de traitement des données météorologiques permettant d'établir le niveau d'humidité des sols superficiels par Météo-France ; ensuite, rendre plus lisibles pour les responsables communaux et les sinistrés les critères mis en oeuvre et, à cet égard, un effort de simplification de leur présentation sera réalisé.

Grand Est suscite la plus grande inquiétude en Moselle. De fait, le 9 décembre 2018, la SNCF a, de son propre chef, modifié le cadencement des TGV reliant Metz à Paris. Les changements d'horaires opérés depuis cette date ont, effectivement, ont, effectivement, été décidés sans concertation aucune avec qui que ce soit. Face aux multiples interrogations suscitées par cette nouvelle politique, la SNCF avance des arguments quelque peu fallacieux. Elle tente, notamment, de faire passer pour des progrès la suppression de trains À cet égard, l'exemple du train de 8h56, qui relie Metz à Paris, est particulièrement parlant. Ce train, l'un des plus utilisés sur ce tronçon, avait purement et simplement disparu de l'offre de la SNCF. Jusqu'à son rétablissement, le 1 avril dernier, les usagers devaient donc se reporter sur le train de 7h26, souvent surbooké ou se rendre à Nancy. Les exemples de changements aberrants sont tout autant parlants dans le sens Paris-Metz, où la SNCF multiplie les Ouigo, qui posent d'autres problèmes. C'est la raison pour laquelle nombre d'élus mosellans élèvent une protestation unanime, soulignant d'une même voix et avec force que tout citoyen est en droit d'attendre qu'un opérateur de services publics prenne des dispositions pour accompagner les usagers et non pour les dissuader en mettant en place des procédures toujours plus complexes. Aussi, madame la secrétaire d'État, pourriez-vous veiller à ce que la SNCF

L'offre Ouigo a été ouverte en juillet 2018 sur cette liaison, avec un aller-retour quotidien, afin d'ouvrir l'accès aux services grande vitesse à des voyageurs très sensibles aux prix. Sur le second semestre 2018, la fréquentation a été particulièrement élevée, avec un total de 120 000 voyageurs transportés. Face à ce succès croissant, SNCF Mobilités a introduit, en décembre 2018, un aller-retour quotidien supplémentaire Ouigo entre Metz et Paris. Pour prendre en considération les critères techniques, économiques et commerciaux spécifiques à Ouigo, le déploiement de ces trains s'accompagne de nécessaires ajustements du plan de transport des TGV classiques, en vue de favoriser un cadencement plus homogène des trains. Je vous indique cependant qu'une attention toute particulière a finalement été portée aux périodes de pointe, avec le maintien systématique de TGV classiques. Depuis le 1 avril 2019, SNCF Mobilités a par ailleurs renforcé la liaison Paris-Metz, avec un aller-retour quotidien supplémentaire en TGV classique. Dans le sens Metz-Paris, vous l'avez dit, SNCF Mobilités a bien positionné un départ TGV classique à 8h56. Dans le sens inverse, deux TGV classiques sont dorénavant proposés en soirée, avec des départs de Paris à 19h40 et 20h48, qui se substituent au train partant à 20h13. Au final, le nouveau plan de transport permet ainsi de proposer un cadencement des TGV de quarante minutes en moyenne durant les périodes de pointe et de deux heures en moyenne pendant les périodes creuses, en laissant le choix entre les offres TGV et Ouigo.

Je tiens à cette occasion à réaffirmer que le Gouvernement est très attaché à ce qu'un dialogue soit ouvert entre SNCF Mobilités et les territoires. La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire crée ainsi, à partir du service annuel 2021, des procédures de consultation et d'information obligatoires

Mizzon, pour la réplique. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d'État, mais je crains fort que la politique menée à l'heure actuelle par la SNCF ne continue à susciter le plus vif mécontentement dans le Grand Est, singulièrement en Moselle, où

les billets sont parmi les plus chers pour la ligne Grand Est et ils s'achètent uniquement internet. En outre, ni les abonnements ni les cartes de réduction SNCF ne sont pris en compte. Il n'est pas non plus possible de réserver une place ou d'acheter un titre de transport

certaines communes ont fait le choix du maintien communal de l'exercice des compétences eau et assainissement entre 2020 et 2026, comme la loi le leur permet. Or, dans le cadre du onzième programme des agences de l'eau, la quasi-totalité des agences ont profité de cette opportunité pour décider d'exclure du système d'aides les communes qui n'ont pas transféré ces compétences à la communauté de communes ou, plus hypocrite, qui n'ont pas de projets intercommunaux. Il s'agit le plus souvent de communes isolées, dont la situation géographique ne rendait pas ce transfert pertinent. En application de la loi du 3 août 2018, les communes qui n'ont pas transféré ces compétences sont dans leur plein droit et n'ont donc nulle raison de s'en trouver pénalisées. Les décisions de ce genre prises par certaines agences de l'eau sont d'autant plus iniques que leurs programmes d'action sont alimentés par des redevances acquittées par tous les usagers de l'eau, même les ruraux. Lors du vote de la loi du 3 août 2018, je déclarais : « Laisser la compétence aux communes qui le désirent est indispensable, mais à condition qu'elles en aient les moyens. [ ...] Sinon, sans moyens financiers, le transfert deviendra obligatoire. » C'est ce que la technostructure est en train de réaliser, car elle n'a pas digéré la dérogation imposée par les représentants du peuple ! Peut-être est-ce d'ailleurs aussi l'occasion de nous interroger sur la raison d'être des agences de bassin, qui ne soutiennent plus les communes, en particulier les plus petites. Elles font partie de ces agences dites « indépendantes » qui coûtent très cher au budget national. Je souhaite donc connaître, madame la secrétaire d'État, les mesures que vous envisagez de mettre en place pour que les agences de l'eau continuent à soutenir financièrement les communes concernées, lesquelles sont bien souvent les plus isolées mais n'ont pas moins besoin que les autres de réaliser des travaux pour distribuer une eau saine à leurs habitants.

la loi du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne remet pas en cause le principe du transfert de ces compétences, prévu notamment par la loi du 7 août 2015 Elle prévoit, vous l'avez dit, d'assouplir la mise en oeuvre de ce transfert, ce qui peut conduire, dans certains cas, à n'opérer le transfert de compétences que le 1 janvier 2026 au plus tard. Il est cohérent que les modalités d'attribution des aides publiques accompagnent ce transfert de compétences. En ce sens, des critères de priorisation et non d'exclusion des dossiers ont été mis en place en octobre 2018 par les comités de bassin, où siègent des élus, dans les onzièmes programmes d'intervention des agences de l'eau, pour accompagner cette structuration des compétences. Les agences font vivre des solidarités : solidarité territoriale entre zones urbaines et zones rurales intercommunale, les EPCI ; solidarité amont-aval à l'échelle du bassin versant et avec les façades littorales en accompagnant les collectivités dans la structuration des compétences eau potable, assainissement et gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, ou Gemapi solidarité internationale en aidant des projets en faveur de pays moins favorisés en matière d'accès à la ressource en eau et d'assainissement. Néanmoins, je vous rassurer en vous disant que les onzièmes programmes n'interdisent aucunement l'attribution de subventions directement aux communes. Celles qui, à ce jour, ont conservé les compétences eau et assainissement ne sont donc pas exclues de tout dispositif d'aides, et ce d'autant moins que la loi du 3 août 2018 permet un transfert progressif de ces compétences vers les EPCI. Il convient enfin de rappeler que ce sont avant tout les communes rurales qui sont éligibles, au titre de la solidarité territoriale, aux aides des agences de l'eau dédiées à l'entretien de leurs réseaux d'eau potable et d'assainissement, et ce indépendamment du transfert de ces compétences aux EPCI.

exemple, la petite commune de Lachapelle-Graillouse doit renouveler ses canalisations d'eau qui datent de 1940. Loire-Bretagne ne finance pas, alors que Rhône-Méditerranée-Corse l'aurait fait. Exactement ! Pas d'aide pour les stations d'épuration inférieures à 180 habitants, comme à Saint-Étienne-de-Lugdarès. Ces Français n'ont pas les mêmes droits que ceux des grandes villes

Ouvrez les yeux ! Il y a deux France : la vôtre, celle des grandes métropoles, et la mienne, celle des ruraux et des oubliés

Madame la secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur le caractère accidentogène du tronçon Saintes-Dompierre-sur-Charente de la route nationale 141. En effet, depuis 2014, on compte 8 décès sur les 9 kilomètres qui composent ce tronçon. À cela s'ajoutent de nombreux blessés et un niveau de dangerosité important pour les quelque 12 000 véhicules qui empruntent quotidiennement cette route nationale. La commune de Chaniers a essayé, à son échelle, de faire face à cette situation en installant deux radars pédagogiques et en transformant le lieu-dit du Maine-Allain en agglomération. Parallèlement et de façon étonnante, une étude récente, conduite dans le cadre de la démarche « sécurité des usagers sur les routes existantes », a indiqué que l'accidentologie de cette zone ne présente pas de caractéristiques importantes d'insécurité, malgré l'avis unanime des élus concernés, malgré les études réalisées par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, ou Cérema, et malgré la sombre réalité des chiffres. Face à cette situation, les élus locaux ont entrepris d'alerter l'ensemble des services de l'État sur l'urgence de la situation. Mais rien n'y fait, les maires des communes concernées n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante. Aussi, madame la secrétaire d'État, je souhaiterais qu'entre les murs de la Haute Assemblée le Gouvernement s'engage à trouver une solution rapide et efficiente, afin que le tronçon Saintes-Dompierre-sur-Charente de la route nationale 141 ne soit plus un lieu de drames humains. Que compte-t-il faire ?

Ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre. Les aménagements de sécurité menés sur le réseau routier national non concédé sont programmés suivant les résultats de la démarche de sûreté des usagers sur les routes existantes. Elle est mise en oeuvre en application des articles L. 118-6 et de l'article réglementaire correspondant du code de la voirie routière, découlant de la mise en oeuvre de la directive relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières. Cette démarche permet de hiérarchiser les enjeux de sécurité à partir de l'analyse systématique des accidents corporels. Sur les sections classées comme prioritaires compte tenu de l'accidentalité constatée, un programme d'actions est alors défini, afin d'améliorer la sécurité de l'itinéraire. Les études effectuées par la direction interdépartementale interdépartementale des routes Atlantique ont révélé qu'il existait une zone d'accumulation d'accidents au niveau de l'intersection entre la RN 141 et la RD 131 sur la commune de Chaniers. À cet effet, l'État a réalisé et financé intégralement, entre 2015 et 2016, l'aménagement d'un carrefour giratoire au niveau de cette intersection, pour un montant de 1 million d'euros. La mise en service de cet aménagement étant relativement récente, il n'est pas possible, à ce stade, de mesurer les effets sur l'accidentalité. On notera néanmoins qu'il n'y a heureusement pas eu de nouvel accident mortel à ce niveau depuis la mise en service du carrefour giratoire. S'agissant plus particulièrement du hameau du Maine-Allain sur la RN 141, les études commandées par la commune de Chaniers auprès du Cérema concluent que les difficultés qui y sont ressenties sont avant tout la conséquence d'absence d'aménagement adapté au contexte urbain. Ce type d'aménagement, en agglomération, relève de la compétence de la collectivité. Je tiens, par ailleurs, à rappeler que l'infrastructure n'est pas le seul facteur d'accidents. La majorité des accidents reste liée au comportement à risque de certains conducteurs. Le dernier accident mortel, survenu en février dernier sur la RN 141, était malheureusement dû à un endormissement. Afin de lutter contre les cas de vitesse excessive pratiquée par certains usagers de la route, il convient d'examiner, en liaison avec le préfet de département, d'autres solutions, tel le renforcement des contrôles de vitesse.

par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, le pôle « monde » du tribunal d'instance de Paris ! Ce délai était de dix-huit mois en 2007 ; on le considérait alors déjà comme anormalement long. Un tel retard trouvait son origine dans la multiplication des demandes injustifiées de CNF. En effet, le nombre de ces demandes était passé, entre 2004 et 2006, de 9 463 à 36 175, sans que les effectifs du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris autant. Grâce à la désignation de dix nouveaux agents ainsi qu'au regroupement géographique de l'ensemble des tribunaux d'instance parisiens, le délai moyen de délivrance des certificats de nationalité française fut alors réduit à douze mois. Comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, ce délai est en moyenne de trente-six mois. L'attention de la direction des services judiciaires a été appelée sur la nécessité de renforcer les moyens humains.

pour les Français nés et établis hors de France. Il conviendrait notamment de mettre en place un système de filtrage des demandes qui n'ont aucune chance de prospérer, car elles sont nombreuses ! Par ailleurs, où en sommes-nous de la numérisation des dossiers ? cas impératif de ramener le délai de délivrance des certificats de nationalité française à douze mois, délai atteint il y a dix ans. La parole

Le pôle de la nationalité du tribunal d'instance de Paris est destinataire des demandes de certificat de nationalité française émanant des personnes domiciliées à l'étranger, ce qui correspond à plus de 30 000 demandes par an ; en deux ans, ce nombre a augmenté Cette augmentation a provoqué, depuis 2005, un doublement du stock des dossiers en cours, et ce en dépit d'un taux de couverture des demandes relativement constant et, depuis le début de l'année 2019, supérieur à 100 %. Des moyens, tant organisationnels qu'humains, ont été déployés pour résorber ce stock et réduire en conséquence le délai de traitement des demandes. Tout d'abord, une rationalisation du traitement des dossiers et,

Ensuite, une priorisation du traitement des demandes a pour objectif d'apporter immédiatement des réponses aux dossiers dont l'instruction est achevée et de compléter l'instruction des demandes fondées sur des motifs permettant de justifier la délivrance d'un certificat de nationalité française. Enfin, une réorganisation du service, visant à l'adapter à ses effectifs actuels et prévisibles, a permis d'entamer le stock des dossiers, de telle sorte qu'une réduction du délai de traitement peut raisonnablement être attendue. le sénateur, que les services du ministère de la justice continueront de porter une attention particulière aux modalités de délivrance de ces documents, qui revêtent une importance particulière pour les personnes qui le sollicitent.

seule à même d'y mettre un terme. En effet, si l'ordre public doit être la règle, la réponse ne saurait être uniquement répressive, d'autant que cette approche a eu des conséquences dramatiques pour nombre de manifestants parfaitement pacifiques.

leurs rideaux baissés. Nous le savons bien, le chiffre d'affaires perdu lors de ces journées, qui devraient être les meilleures du point de vue commercial, ne se rattrape jamais. Au fil du temps, le comportement des consommateurs évolue : ils choisissent d'aller dans les centres commerciaux de périphérie, ou de commander par internet, pour ne pas se trouver en ville au moment des manifestations. Dès lors, l'attractivité future de nos centres-villes est gravement menacée et doit faire l'objet de toute l'attention de l'État comme des collectivités. Quant au fonds de 3 millions d'euros envisagé par le Premier ministre pour des opérations de promotion commerciale, il n'est pas à l'échelle de la problématique. Concernant le soutien aux commerçants indépendants eux-mêmes, la réponse du Gouvernement est là aussi trop limitée, dans le temps comme dans ses effets, car l'étalement de la dette, qu'elle soit fiscale ou sociale, n'apporte aux entreprises qu'une solution de court terme. Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances avait, en son temps, ouvert la voie à une possibilité d'exonérations de taxes et cotisations sociales. Pouvez-vous nous dire, monsieur le secrétaire d'État, le nombre d'exonérations accordées à ce jour et leur montant total ? La grande absente des mesures annoncées par le Gouvernement reste la question de la dégradation de la trésorerie de ces sociétés ; on sait qu'elle préfigure souvent des redressements ou des liquidations. En la matière, vos appels incantatoires à la plus haute bienveillance des banques risquent d'être insuffisants. Sur un autre plan, on entend que les compagnies d'assurance réfléchiraient à demander, à l'avenir, une surprime aux établissements commerciaux de centres-villes, ce qui reviendrait pour ceux-ci à subir une triple peine : réparations, perte de chiffre d'affaires, augmentation des primes d'assurance. Alors, même si ce gouvernement, depuis vingt et une semaines, ne parvient pas à trouver de sortie à la crise politique, peut-être peut-il répondre aux attentes de nos concitoyens artisans et commerçants indépendants, qui, au fond, en paieront très largement la note

Permettez-moi, avant de répondre à votre question relative aux modalités d'intervention du Gouvernement, de souligner que cet impact recouvre, évidemment, les charges liées à des sinistres ou à des dégradations,

La réponse du Gouvernement s'est faite en trois temps. Dès le mois de novembre 2018, c'est-à-dire dès les premiers jours de la mobilisation, nous avons demandé à l'ensemble de nos services d'être extrêmement bienveillants envers les commerçants et les chefs d'entreprises concernés, notamment par l'octroi de délais de paiement. Cela s'est fait dans le cadre d'une relation bilatérale assez informelle, mais courante en la matière, et nous avons veillé à ce que l'ensemble de nos services appliquent ces instructions.

Monsieur le secrétaire d'État, en France, la loi donne le statut de service public au transport par remontées mécaniques, y compris pour les remontées à vocation touristique dans le contexte concurrentiel des stations. Ce choix singulier, que la France est seule à avoir fait parmi ses concurrents dans l'arc alpin, comporte des limites dont il est de plus en plus difficile de s'accommoder sans nuire à l'économie de nos stations. L'application que nous avons ainsi faite des délégations de service public à l'économie très particulière des domaines skiables est une construction juridiquement instable,

Dans ce cas d'espèce, une convention « loi Montagne » avait été rédigée entre la collectivité et l'opérateur privé historique de la station, propriétaire des remontées mécaniques, des autres biens et du foncier. Arrivés au terme du contrat, délégant et délégataire ont appliqué les clauses de rachat prévues au contrat, mais se sont heurtés au contrôle de légalité : ces clauses ont été jugées illégales, alors même qu'elles avaient été rédigées et validées par les conseils juridiques et l'administration. Depuis l'arrêt du Conseil d'État du 21 décembre 2012, on savait que les clauses d'indemnisation des biens de retour fixées à des valeurs supérieures à la valeur nette comptable étaient regardées comme non conformes, ce qui pose un problème partout où de telles clauses ont été conclues. L'arrêt va plus loin : il fait craindre que ces clauses soient inopérantes en pratique, ce qui modifie l'équilibre économique du contrat.

arrêt constitue un revirement jurisprudentiel, qui affecte, directement ou indirectement, toutes les concessions de remontées mécaniques. L'impermanence des règles pose un problème de loyauté, dès lors qu'on applique la nouvelle règle à des contrats signés antérieurement à l'arrêt. C'est encore C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'exploitants qui étaient propriétaires d'une exploitation antérieurement à leur premier conventionnement et que tout le monde- tant leurs conseillers juridiques que les administrations -poussait à signer des clauses d'indemnisation, jugées illégales trente ans plus tard. Outre les contentieux qui ne manqueront pas de naître de cette situation invraisemblable, ces changements incessants sont de nature à détourner les investisseurs privés des domaines skiables. Une telle situation n'est bonne ni pour les délégants ni pour les délégataires. Conscients des difficultés nées de l'application du régime des délégations de service public aux remontées mécaniques, Domaines skiables de France et l'Association nationale des maires des stations de montagne se sont réunis plusieurs fois dans le but de formuler des propositions communes. Dans l'hypothèse où les évolutions du droit rendraient caduques des dispositions contractuelles conclues antérieurement, l'équilibre économique du contrat doit être maintenu. Ma question, monsieur le secrétaire d'État, est donc la suivante : comment comptez-vous sécuriser le classement des biens et leur indemnisation tel que stipulé dans les contrats conclus antérieurement aux évolutions du droit ? La parole

Il résulte des articles L. 342-9 et suivants du code du tourisme que les communes, leurs groupements et les départements sont compétents pour les services de remontée mécanique, qu'ils peuvent assurer soit directement, en régie simple ou personnalisée, soit indirectement, à l'aide d'une délégation de service public. Dans cette seconde hypothèse, l'autorité concédante et son cocontractant sont soumis au régime des biens de retour, tel que cela a été établi par le Conseil d'État. Dans une décision du 21 décembre 2012,, que vous avez citée, le Conseil a estimé que « l'ensemble des biens meubles ou immeubles, nécessaires au fonctionnement du service public », dont la convention a mis « à la charge du cocontractant les investissements correspondants à la création ou à l'acquisition » constituent une catégorie de biens qui font retour gratuitement à l'autorité concédante à l'issue de la convention.

Cette solution est justifiée par le fait que les biens ainsi acquis ont fait l'objet d'une rétribution au concessionnaire. En effet, d'une part, le concessionnaire peut amortir le coût de ces équipements pendant la durée de la concession, à l'aide du prix payé par les usagers du service ; d'autre part, et à défaut, l'autorité concédante lui doit une indemnité lorsque les biens ne peuvent être amortis, si la durée de la concession est inférieure à celle de l'amortissement, que cela soit décidé ou que la concession ait été résiliée de manière anticipée, pour faute du cocontractant ou pour motif d'intérêt général. S'agissant de l'application de ce régime à la situation des concessionnaires de remontées mécaniques qui étaient propriétaires de leurs équipements avant la loi Montagne du 9 janvier 1985, ceux-ci disposaient d'une période transitoire de quatorze ans pour faire le choix soit de la cession onéreuse de leur équipement à la collectivité compétente, soit du régime conventionnel. Pour ceux qui ont choisi la seconde option, il n'est pas douteux que l'apport des équipements par le concessionnaire a été pris en compte au stade de la négociation du contrat. Dans le cas contraire, et si la situation aboutit à un déséquilibre contractuel, que le consentement du concessionnaire a été vicié, ou bien qu'une évaluation erronée des biens apportés a été faite de bonne foi, alors le concessionnaire est fondé à faire valoir ses droits à indemnité. Telles sont les précisions que je pouvais vous apporter, monsieur le sénateur.

Oui, un fait colonial, je persiste et je signe ! Je m'explique : non seulement ce foncier continue d'appartenir, pour 95 %, à l'État, fait unique dans toute la France, mais surtout il est géré de façon jalouse et stérile, comme le dénonçait le Sénat dans un rapport de 2015 : l'État fait fi de ses obligations, malgré les exigences de la loi.

ce texte, dispose : « Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'évaluation cadastrale des parcelles de forêt exploitées, concédées ou gérées par l'Office national des forêts

est redevable de cette taxe sur les parties du domaine forestier qu'il exploite et dont le produit des ventes de bois et concessions est affecté à son budget. Pourtant, à ce jour, soit vingt-quatre mois après la promulgation de la loi, rien n'a été fait La perception de la taxe n'a toujours pas lieu ; c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui échappent ainsi aux collectivités de Guyane, dont bon nombre sont déjà exsangues financièrement. J'ai interpellé le directeur régional des finances publiques de Guyane sur ce sujet, à la suite d'une lettre ouverte d'un agent de son administration se disant sanctionné pour avoir voulu lancer la procédure de recouvrement de cette taxe. Monsieur le secrétaire d'État, ma question est simple : qu'en est-il ? Qu'attend le Gouvernement pour assumer ses responsabilités et demander à l'ONF de payer ce qu'il doit aux collectivités ?

Soyez assuré, monsieur le sénateur, que ce sujet retient toute l'attention du Gouvernement et, en particulier, celle de nos services. Comme vous le savez, ce dossier est extrêmement complexe, du fait de l'étendue de la forêt amazonienne guyanaise et des caractéristiques de cette dernière, très différentes de celles des bois et forêts métropolitains. Aussi, nos services, en association avec ceux du ministère de l'agriculture, travaillent sur une taxation prenant en compte les spécificités de la forêt amazonienne de la Guyane et, en particulier, sa surface, qui s'élève à 5 millions d'hectares, contre 11,7 millions d'hectares de forêts dans tout l'Hexagone, ainsi que sa rentabilité réelle. Je vous confirme qu'il sera bien procédé à l'émission d'une taxation des parcelles gérées par l'ONF au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2018, d'ici à la fin de l'année 2019, conformément aux dispositions évoquées, que vous aviez défendues dans cet hémicycle.

conformément à ce qui a pu être fait en France et dans d'autres territoires outre-mer, le foncier de la Guyane revienne aux Guyanais, dans le cadre d'un transfert de compétences. La

attachent une haute importance à la réalisation de ce projet. Conscients de son importance stratégique, ils ont, depuis leur arrivée en fonction, consacré une grande part de leur énergie à la recherche de financements innovants et spécifiques. Un projet de cette ampleur implique, comme vous l'avez fait remarquer, la concordance de plusieurs sources de financement. Ce sera le cas pour le canal Seine-Nord Europe, dont le coût total serait, ainsi que l'a rappelé le Président de la République, réparti entre 2 milliards d'euros de subventions européennes, 1 milliard d'euros de ressources propres des collectivités, la mise en place par l'État de taxes nationales à assise locale qui permettront de gager un emprunt d'1 milliard d'euros, ainsi que 700 à 900 millions d'euros issus d'un emprunt garanti par la Société du canal Seine-Nord Europe, devenue régionale. Vous m'interrogez plus particulièrement sur la part de ce financement revenant à l'État. Elle doit, comme vous le savez, intervenir au 1 janvier 2021. Sachez, monsieur le sénateur, que ce délai est utilement mis à profit par le Gouvernement et que, contrairement à ce que vous pouvez craindre, l'État ne se désengage pas ; bien au contraire, il fait des propositions et cherche les bonnes solutions. Nous avons notamment suggéré l'instauration d'une taxe spécifique à la région des Hauts-de-France, même si cette solution semble juridiquement fragile d'après l'avis qu'a récemment rendu le Conseil d'État. D'autres pistes sont à l'étude, mais elles nécessitent des analyses juridiques approfondies et, pour certaines d'entre elles, des échanges avec la Commission européenne afin de bien cerner ce que permet le cadre européen. Vous évoquez une troisième piste : l'inscription de crédits budgétaires dédiés. Le Gouvernement considère que cette solution ne devra être retenue qu'en dernier recours, dans la mesure où elle ne permet pas d'associer les futurs bénéficiaires du canal à son financement.

Comme vous le savez, tel est l'objet de l'article 36 du projet de loi d'orientations des mobilités, qui prévoit, d'une part, de ratifier l'ordonnance du 21 avril 2016 relative à la Société du canal Seine-Nord Europe, et, d'autre part, d'autoriser le Gouvernement à prendre, par la voie d'une nouvelle ordonnance, des dispositions visant à la transformation de cet établissement public national en établissement public local. Soyez assuré, en tout état de cause, monsieur le sénateur, que le Gouvernement est déterminé à faire aboutir ce projet

Or, à Wallis-et-Futuna, les missions de la police aux frontières sont actuellement assurées par la gendarmerie, et ce sans aucune base juridique. Plus précisément, jusqu'à l'installation des gendarmes mobiles sur le territoire, la police aux frontières était assurée par quatre gardes territoriaux, sous la responsabilité d'un gendarme référent. Depuis leur installation, les gendarmes mobiles ont repris le service, mais ils continuent à faire appel aux gardes territoriaux lorsqu'ils rencontrent des problèmes d'effectifs. se fait, bien sûr, sans habilitation officielle ni base normative. Cette situation bancale ne saurait perdurer. Je sais que plusieurs pistes sont à l'étude. pour des raisons budgétaires, chaque service se renvoie la balle, si je puis dire, entre la direction centrale de la police aux frontières, la direction des douanes et la gendarmerie. Monsieur le secrétaire d'État, la meilleure piste ne serait-elle pas une collaboration avec la police aux frontières de Nouvelle-Calédonie, qui formerait les gardes territoriaux de Wallis-et-Futuna et collaborerait avec eux ? La surveillance aux frontières est un métier de policier, et non pas une mission de douanier. Je souhaiterais donc savoir ce que compte faire le Gouvernement pour mettre en place une solution plus viable et officielle, afin d'assurer cette prérogative régalienne. La

la direction centrale de la police aux frontières et la direction de la gendarmerie nationale, réflexion qui associera aussi la direction de la douane, afin de mettre en place un système qui soit, comme vous le souhaitez, plus efficace et conforme à la réglementation. Je ne manquerai pas de porter personnellement auprès de Laurent Nunez et de Christophe Castaner votre message

reçoit parfois le renfort de la garde territoriale. Face à cette situation qui n'est pas pleinement satisfaisante, nous sommes à l'heure des réflexions. Vous avez d'ailleurs vous-même mis une piste sur la table ce matin, et je m'en ferai l'écho auprès de mes collègues pour

Les entreprises de réservation en ligne, comme Airbnb, Booking.com, Expedia Group ou TripAdvisor, contribuent à des violations de droits humains des Palestiniens, en proposant plusieurs centaines d'hébergements et activités dans les colonies illégales de peuplement israéliennes en territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est.

2019 intitulé, ces entreprises du numérique induisent en erreur leurs clients, en s'abstenant d'indiquer systématiquement que les offres concernées sont situées dans les territoires occupés. Or, en favorisant l'industrie du tourisme dans les colonies et, en conséquence, l'essor économique de ces implantations qui sont contraires au droit international, Airbnb, Booking.com, Expedia Group et TripAdvisor contribuent au maintien, au développement et à l'extension des colonies de peuplement illégales et en

qui fournissent des informations trompeuses, en s'abstenant d'indiquer que les hébergements proposés sont situés en territoires palestiniens occupés dans des colonies illégales au regard du droit international, et non en Israël.

condamne régulièrement les annonces de construction de nouveaux logements dans les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ainsi que les démolitions et les évacuations forcées en zone C, qui participent de la même stratégie. De même, nous appelons publiquement les autorités israéliennes à reconsidérer ces décisions et à abandonner cette stratégie de colonisation afin de préserver la solution des deux États avec Jérusalem comme capitale. Nous avons tiré les conséquences de cette

informer nos compatriotes des risques encourus lors de séjours à l'étranger et à les sensibiliser sur les mesures et comportements à adopter pour réaliser leurs déplacements dans les meilleures conditions,

Monsieur le secrétaire d'État, lors de mes déplacements en circonscription, je note partout l'inquiétude grandissante de nos compatriotes et de nos conseillers consulaires quant au devenir des postes diplomatiques. Pour répondre à la demande inédite de réduction de 10 % de la masse salariale de la représentation française à l'étranger, les fermetures de certains services et la diminution du personnel ne peuvent être que drastiques. Elles vont toucher directement plus de trois millions de nos concitoyens résidant à l'étranger, mais aussi quelques centaines de milliers de transfrontaliers et les millions de touristes français. Tous les postes sont concernés et nos ambassadeurs, immédiatement sollicités pour faire connaître les économies qu'ils pouvaient réaliser, ont tous fait des propositions, que pour l'instant Je voudrais prendre comme exemple notre poste au Luxembourg, que je connais bien et qui rassemble un certain nombre de problématiques. La population française a dépassé 53 000 résidents- c'est le nombre recensé par les autorités locales -, dont 36 000 inscrits au consulat. Les Français établis au Luxembourg représentent la dixième communauté française dans le monde, à laquelle je me dois d'ajouter les 100 000 frontaliers qui, chaque jour, viennent travailler dans ce pays. Beaucoup préfèrent s'adresser au consulat pour la délivrance de leurs papiers d'identité c'est plus facile pour eux, car ils sont sur place et ne doivent pas prendre deux jours de congé pour effectuer les mêmes démarches dans leur commune. Depuis plusieurs mois, le personnel est soumis à une continuelle pression de la part des usagers mécontents de la diminution des services. Pourtant, les agents ne chôment pas, avec en moyenne trente-six rendez-vous par jour ouvré. Aujourd'hui, nos concitoyens craignent une éventuelle fermeture du consulat, alors même que certains services ne peuvent pas être supprimés- c'est le cas pour les dossiers de nationalité et de bourses scolaires. D'ici à 2020, les services de l'état civil vont être transférés à Nantes. Il semblerait que l'on envisage également de demander à nos concitoyens du Luxembourg de se déplacer à Bruxelles pour certaines démarches administratives ou même de se rendre en France. Or je ne pense pas qu'il soit envisagé d'augmenter le personnel dans les départements frontaliers ou au consulat à à Bruxelles. Monsieur le secrétaire d'État, au vu du nombre important de personnes concernées, pouvez-vous me donner une réponse claire et précise sur les décisions que vous entendez prendre concernant ce poste et, plus généralement, sur les grandes orientations pour l'ensemble du réseau ?

la capacité, pour les Français établis hors de France, d'avoir accès, dans de bonnes conditions, à tous ces services. Cette réorganisation

Ce fonds a vocation à soutenir des actions menées par les pays de l'Union européenne pour apporter une assistance matérielle aux plus précaires. Il permet aux associations françaises de disposer de 100 à 120 tonnes de produits de base, soit près de 30 % des produits distribués dans leurs permanences. Comme vous le voyez, cet apport est essentiel pour assurer une stabilité et une régularité des denrées distribuées aux personnes dans le besoin. Or les représentants de ces associations constatent depuis plusieurs années des retards récurrents de plusieurs mois dans la livraison des produits issus du FEAD. FEAD. Surtout, ils craignent une diminution des moyens alloués dans les années qui viennent. En effet, dans le cadre de la prochaine programmation budgétaire, un changement total de paradigme nous passerions d'un fonds spécifiquement dédié à un pourcentage minimum réservé au sein d'un programme global, le FSE+, laissant la possibilité aux États membres, s'ils le souhaitent, de consacrer une enveloppe plus importante à l'aide aux plus démunis.

Les échanges entre le Président de la République et les élus locaux ont montré l'importance de ce sujet, qui induit un sentiment de dépossession progressive des communes rurales de leurs missions essentielles. Les élus aimeraient qu'au minimum chaque intercommunalité dispose de la capacité de délivrer les cartes nationales d'identité. Le Président de la République s'est engagé, lors du débat qui s'est tenu le 15 janvier au Grand Bourgtheroulde, à « rouvrir le sujet pour les cartes d'identité, les passeports et les permis de conduire ». Le grand débat étant terminé, je souhaiterais connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet et, au-delà, sur les mesures qu'il compte prendre pour conforter les communes et redonner confiance et espoir aux maires. À cet égard, permettez-moi de vous rappeler que les maires aspirent notamment à un allégement des normes, à une visibilité sur l'évolution de leurs ressources, à un meilleur fonctionnement des intercommunalités ou encore à une amélioration de leur statut.

le cadre du programme Action publique 2022, un plan social de grande ampleur est prévu chez Atout France. Au-delà de la préoccupation légitime des salariés de l'agence, nous sommes nombreux à nous interroger sur le choix stratégique du Gouvernement, qui a pour objectif d'accueillir 100 millions de touristes d'ici à 2020, mais cela, si l'on comprend bien, avec des moyens et des effectifs en baisse Vouloir économiser 4 millions d'euros, alors que l'action d'Atout France sur notre rayonnement à l'étranger est majeure, est plus que surprenant. La filière du tourisme représente des centaines de milliers d'emplois en France. Cette richesse contribue largement à notre croissance et à un rayonnement culturel qui va bien au-delà du simple secteur touristique.

nous aurions très prochainement à mener une réflexion stratégique sur la promotion touristique. Il est inutile de vous dire que les acteurs du tourisme, notamment Atout France, attendent avec impatience l'issue de cette réflexion.

des solidarités et de la santé. Monsieur le secrétaire d'État, ma question s'adressait à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Les compléments alimentaires sont des denrées dont le but est de compléter un régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Ils sont conditionnés sous forme de comprimés, de gélules, de pastilles ou encore d'ampoules et peuvent contenir des vitamines et minéraux, des plantes ou d'autres ingrédients à but nutritionnel ou physiologique. La fabrication et la commercialisation des compléments alimentaires sont soumises à une réglementation européenne. N'étant pas des médicaments, ils sont ensuite vendus sans ordonnance et largement distribués dans les pharmacies, les grandes surfaces, les magasins spécialisés ou sur internet. Il faut à cet égard rappeler que, mal utilisés, ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs et entraîner des effets toxiques, en raison notamment de surdosage ou de surconsommation du fait de la prise concomitante de plusieurs types de produits. En outre, les compléments alimentaires sont souvent prescrits aux personnes âgées souffrant de dénutrition. Certains facteurs tels que la perte de mobilité, combinés à l'augmentation des besoins métaboliques liés à l'âge, peuvent en effet nécessiter une supplémentation, parallèlement au maintien d'une alimentation équilibrée.

m'indiquer, monsieur le secrétaire d'État, quelles sont les modalités de prescription de ces compléments alimentaires, ainsi que leurs conditions de prise en charge par la sécurité sociale ? Existe-t-il des recommandations ou un guide de bonnes pratiques en la matière ? ? Plus précisément, des réflexions sont-elles en cours sur un éventuel encadrement de ces prescriptions et sur une plus grande transparence des frais qu'elles engendrent ? Je vous remercie de votre éclairage.

aura permis d'en parler dans cet hémicycle. Elle constitue un obstacle à une prise en charge précoce. En France, en 2018, la prévalence de la dénutrition demeurait élevée. On estime en effet à 2 millions le le nombre d'individus qui en souffrent. Cette prévalence augmente avec l'avancée en âge et touche par conséquent davantage les personnes âgées, comme vous l'avez indiqué. En raison de l'évolution démographique de la population et de l'augmentation des pathologies chroniques, une augmentation importante du nombre de personnes touchées est ainsi à redouter dans les prochaines années. Nous savons ce qui ce qui attend notre pays ... Les conséquences de la dénutrition sont multiples. C'est un facteur majeur de la perte d'autonomie à l'origine de chutes, d'un état dépressif, d'une altération de la qualité de vie en général et, surtout, de la pérennisation d'un déséquilibre alimentaire aggravant aggravant une dénutrition déjà existante. Vous m'interrogez plus spécifiquement sur la prescription des compléments alimentaires. Vous le savez, ces compléments alimentaires sont classés, conformément à la réglementation européenne, comme des denrées alimentaires et ne font pas l'objet d'une prescription médicale en tant que telle. Toutefois, le ministère chargé de la santé recommande de consulter un médecin avant tout achat, compte tenu notamment de certaines interférences possibles avec les médicaments que la personne peut prendre en en parallèle. Les compléments nutritionnels oraux sont des mélanges nutritifs complets auxquels il est possible de recourir dans le cadre de la stratégie nutritionnelle de la personne âgée. Ils sont prescrits à cet égard par un médecin, à des fins médicales, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé, afin d'augmenter l'apport énergétique et protidique des patients dénutris. Ces produits prescrits, dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste des produits et des prestations remboursables, sont pris en charge par l'assurance maladie.

Le Centre hospitalier du Forez, le CHF, a été créé en 2013 par la fusion des centres hospitaliers de Feurs et de Montbrison. Il est désormais le seul hôpital public de l'arrondissement de Montbrison, territoire qui compte plus de 180 000 habitants. À la suite de cette fusion, plusieurs activités ont fermé ou ont été regroupées sur un seul site. Quant aux effectifs, ils ont été réduits. Alors qu'il connaissait des excédents budgétaires avant la fusion, le CHF est désormais en déficit chronique. Cela n'a rien d'étonnant, car, avec le système de tarification à l'activité, la suppression de services entraîne, de fait, la réduction des recettes. de janvier dernier, les membres du conseil de surveillance du CHF ont ouvert la voie à un nouveau recul de l'offre publique de soins : ils ont ainsi acté le principe du transfert à un nouveau gestionnaire de l'autorisation d'exploiter l'Ehpad du Centre hospitalier qui n'a jamais été suggérée dans le projet médical, semble exclusivement motivée par la nécessité de faire face à la mise aux normes de cet établissement de 209 lits, laquelle est devenue indispensable. L'hypothèse d'une rénovation sur le site actuel semble à ce jour écartée. Elle aurait pourtant un pourtant un double intérêt : elle serait moins coûteuse et permettrait de conserver l'Ehpad en centre-ville, situation plus propice à la mixité intergénérationnelle. L'hypothèse envisagée actuellement de reconstruire le centre sur un autre site serait plus onéreuse

entre les deux sites, elle n'a pu l'enrayer dans la durée, la difficulté majeure de recrutement médical ayant contraint l'établissement à adapter son organisation, voire à renoncer à certaines activités.

l'établissement et le conseil départemental -, de la nécessité d'améliorer les conditions d'accueil des personnes âgées qui y sont prises en charge en engageant un projet d'investissement. Cependant, la situation financière générale du Centre hospitalier du Forez, malgré le soutien important de l'ARS, ne l'autorisant pas à contracter les nouveaux emprunts nécessaires

Il revient au conseil de surveillance de l'établissement de se positionner sur les modalités de mise en oeuvre de ce transfert. Dans ce cadre, l'établissement explore différentes hypothèses visant à garantir à la fois l'accessibilité financière du nouvel établissement par un reste à charge comparable à ceux des Ehpad publics du département de la Loire, la poursuite par le nouvel établissement de son rôle naturel d'aval du Centre hospitalier du Forez en matière de gériatrie, et la possibilité pour les personnels de l'Ehpad de poursuivre leur mission sous le statut de la fonction publique hospitalière.

d'État, j'évoquerai ce matin la nécessité d'une meilleure adéquation entre les indicateurs administratifs et la prise en charge sanitaire dans les Hauts-de-France. J'attire l'attention du Gouvernement sur le zonage des médecins généralistes publié en décembre 2018, selon une nouvelle cartographie des zones d'intervention prioritaire, les ZIP, et des zones d'action Vous le savez, les ZIP ouvrent droit pour les médecins aux aides à l'installation de l'assurance maladie de l'État et aux exonérations fiscales au titre de la permanence des soins ambulatoires. Les ZAC ouvrent droit aux seules aides de l'État. La détermination de ces zonages est maintenant nationale. Or l'État a fixé, pour les Hauts-de-France, les seuils d'intervention à 8,3 % de la population pour les ZIP, quand le taux national est de 18 %, et à 38,4 % de la population pour les ZAC, quand le taux national est de 56 %. Ces taux pour le moins très inférieurs aux taux nationaux devraient susciter une réflexion sur la prise en charge sanitaire. Cette nouvelle cartographie fait de la région des Hauts-de-France la troisième région la moins bien dotée de ces dispositifs, bien loin de la réalité des indicateurs de santé fortement dégradés. En effet, dans les Hauts-de-France, la mortalité générale est supérieure de 20 % à la moyenne nationale. Quant à la surmortalité des moins de 65 ans- soit la mortalité prématurée -, elle est supérieure de 33 % pour les hommes et de 26 % pour les femmes aux moyennes nationales.

et de la précarité, les leviers pour agir sur le zonage des médecins généralistes, maillons essentiels de la prise en charge sanitaire, devraient être revus pour favoriser une installation territorialisée cohérente avec le besoin du territoire régional. Quelles mesures concrètes envisagez-vous de prendre pour améliorer la situation dans les Hauts-de-France, et dans quels délais ?

où sont mobilisées les aides à l'installation et au maintien des médecins. L'agence régionale de santé Hauts-de-France a ainsi révisé son zonage à la fin de l'année 2018. L'objectif, partagé, est de favoriser une meilleure répartition des professionnels sur le territoire. L'indicateur pour la détermination des zones est l'accessibilité potentielle localisée, l'APL, à un médecin. Elle intègre le nombre de médecins généralistes, leur activité, le temps d'accès au praticien et le recours aux soins des habitants par classes d'âge. Cet indicateur, dont les acteurs les acteurs saluent la construction robuste, objective la situation de chaque région en termes d'accès à un médecin. La méthodologie prévoit que les agences régionales de santé peuvent utiliser des indicateurs complémentaires pour apprécier les problématiques locales, comme l'état de santé de la population. Une

Les ARS ont donc déterminé les zones prioritaires éligibles à toutes les aides, ainsi que des zones complémentaires éligibles aux aides régionales et locales. La rénovation du zonage a permis un élargissement des territoires éligibles et un soutien financier plus important sur l'ensemble du territoire.

Grâce aux critères objectifs et aux multiples adaptations possibles, l'ARS Hauts-de-France a déterminé les zones en tension tout en portant une attention particulière à l'état de santé de la population et aux territoires défavorisés d'un point de vue social. Par ailleurs, les zones non retenues au sein du zonage peuvent bénéficier d'autres mesures d'accompagnement à l'échelon local. Enfin, la réglementation prévoit une révision de l'arrêté régional définissant le zonage tous les trois ans. Une modification du zonage est possible en tant que de besoin pour tenir compte d'une éventuelle évolution de l'offre durant la période. Ce dispositif de zonage est construit de telle sorte

ma question s'adressait à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Elle porte sur l'avenir de la maternité du Centre hospitalier René-Pleven à Dinan. Appartenant au territoire de santé Saint-Malo-Dinan, qui couvre 138 communes pour 264 000 habitants, soit 8 % de la population bretonne, sur l'est des Côtes-d'Armor et le nord de l'Ille-et-Vilaine, l'hôpital de Dinan fait partie, depuis 2011, de la communauté hospitalière de territoire Rance Émeraude. Avec une capacité de 603 lits, l'hôpital de Dinan est un établissement de proximité centré sur les activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et de prise en charge des personnes âgées. Il compte 7 plateaux techniques. Un projet de fusion des 3 centres hospitaliers de Dinan, de Cancale et de Saint-Malo est en cours d'élaboration à la demande de l'ARS Bretagne. Cette fusion devrait officiellement voir le jour au 1janvier 2020. À l'occasion de la cérémonie des voeux au personnel hospitalier en janvier 2019, la chef de service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de Saint-Malo a mis le feu aux poudres en déclarant que cette fusion ne pourrait avoir lieu

Le territoire de santé a enregistré 2 457 naissances en 2017, dont près de 700 dans la seule maternité de Dinan, contre 778 en 2014. Certes, seules 59 % des parturientes du bassin de vie de Dinan accouchent à la maternité de Dinan, mais des marges de manoeuvre existent pour faire augmenter ce taux, notamment en proposant des services complémentaires comme l'accouchement naturel. Par ailleurs, si la situation financière de l'hôpital de Dinan est assez difficile-

ont été conduits en partenariat avec l'ARS. Il semble par ailleurs que l'ARS soutienne le maintien de la maternité de Dinan et qu'elle souhaite que des investissements soient réalisés pour renforcer l'attractivité de la maternité. Monsieur le secrétaire d'État, il est indispensable de rassurer les personnels et la communauté médicale de l'hôpital de Dinan, la population, ainsi que les élus locaux : quel est l'avenir de la maternité de Dinan ?

des établissements, afin de renforcer la démographie médicale et de permettre une répartition et une graduation des soins adaptées aux besoins du territoire et de ses populations.

respectivement maires des trois communes, avec la direction du GHT et les trois présidentes des commissions médicales d'établissement, a décidé d'acter cette fusion, qui doit s'appuyer sur la construction d'un projet médical partagé. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une situation financière du Centre hospitalier de Dinan effectivement dégradée, vous l'avez rappelé, et doit permettre de développer son activité. Concernant la filière périnatalité, le projet médical partagé du Groupement hospitalier de territoire Rance Émeraude,

des accouchements réalisés sur le territoire concerné. Le projet de territoire vise ainsi à conforter l'image de la maternité de Dinan, qui dispose d'un véritable potentiel de développement, et à donner plus de visibilité aux futurs parents sur l'offre proposée par l'établissement. La parole

Monsieur le secrétaire d'État, alors que la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a apporté des améliorations sensibles pour la prise en charge de nos aînés dépendants à domicile, le sujet de la prise en charge en établissement reste pendant. Lorsque le maintien chez soi a atteint ses limites, les familles sont trop souvent, hélas ! confrontées à la difficulté de trouver une place en Ehpad. Aussi aimerais-je savoir quels moyens le Gouvernement entend dégager afin d'autoriser la création de places supplémentaires dans ces établissements, singulièrement dans les territoires tels que mon département de la Haute-Vienne, où les besoins sont les plus criants au regard de la pyramide des âges, et ce afin d'accueillir convenablement les personnes âgées en situation de grande dépendance qui ne

en 2050, on le sait, car cela suscite un certain nombre de débats, près de 5 millions de Français auront plus de 85 ans, soit trois fois plus qu'aujourd'hui. Le nombre d'aînés en perte d'autonomie aura pour ainsi dire doublé.

la question du nombre de places en Ehpad et de leur accessibilité, mais la difficulté est aussi, et parfois surtout, celle du coût de l'entrée en Ehpad pour les personnes, cette question renvoyant à celle des financements publics apportés aux Ehpad comme aux personnes âgées. Dans son rapport, Dominique Libault aborde dans le détail ces questions et formule des propositions propositions ambitieuses. Des mesures fortes ont également été engagées dès 2018, je le rappelle, avec une feuille de route destinée à répondre très vite à l'urgence qui s'exprimait dans ces établissements. Les principales mesures de cette feuille de route portaient bien entendu sur le financement des Ehpad : moratoire dans la mise en oeuvre de la convergence du tarif dépendance, accélération de la convergence sur le tarif soins pour permettre aux établissements de recruter plus de personnels soignants. Aujourd'hui, sur la base des propositions de Dominique Libault, nous devons répondre à un double enjeu d'accessibilité et d'hétérogénéité de l'offre, à domicile comme en établissement. C'est donc à une réelle transformation de l'offre entre domicile et Ehpad que nous devons nous atteler, pour trouver la solution la plus adaptée aux besoins et aux budgets de chacun de nos aînés. Pour cela, des mesures structurantes devront être prises dans une grande loi, laquelle sera présentée en conseil des ministres à l'automne,

la réalité, c'est que, actuellement, les demandes de création de places portées par les conseils départementaux se heurtent très souvent- trop souvent ! -au refus des ARS, qui ne disposent pas ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour autoriser la création de lits. Les listes d'attente s'allongent et les familles sont dans le plus grand désarroi. Nous pouvons tous ici en témoigner, nous en recevons régulièrement. Si le sujet du coût du reste à charge, vous l'avez évoqué, est explosif, celui des délais d'attente avant d'obtenir une place en établissement ne l'est pas moins. Les deux appellent conjointement une réponse rapide sur les moyens précis, car c'est bien une question de moyens financiers,

apporte des solutions pérennes pour que les familles ne soient pas pénalisées par une double peine : la difficulté à trouver une place, celle ensuite à faire face financièrement. C'est toute la question de la solidarité et de la prise en charge de la solidarité

Ces baisses importantes de personnels et leurs conséquences sur la prise en charge des patients ont conduit à la démission de l'ensemble du conseil d'administration de cette antenne du réseau ADMR le 9 février dernier. Celle-ci est, dans l'attente, gérée par sa fédération départementale, mais le problème du recrutement reste intact. En premier lieu, ces départs s'expliquent notamment par le planning à la minute, source de beaucoup de stress et de précipitation. Parallèlement, la rémunération n'est pas attractive, alors même que ces professionnels ont de lourdes responsabilités. En Savoie, particulièrement en Tarentaise, la question de la rémunération est d'autant plus primordiale que le coût de la vie en station est important, mais également car cette vallée connaît une situation de quasi-plein emploi. lieu, et cela constitue un élément majeur, le montant des frais kilométriques n'est pas adapté à nos zones montagneuses où les déplacements se comptent en temps et non en kilomètres, d'autant que ceux-ci ne sont désormais plus pris en compte pour les trajets retours. Alors que les Ehpad sont surchargés, qu'il est indispensable de garder nos personnes âgées le plus longtemps possible dans leur environnement familial, que les classes de formation ouvertes n'arrivent plus à être remplies, il devient plus qu'urgent de reconsidérer le mode de recrutement, la rémunération et les conditions de travail des auxiliaires de vie.

Agnès Buzyn avait ainsi annoncé, le 30 mai 2018, lors de la présentation de la feuille de route pour les personnes âgées, une refonte du système de financement des services à domicile.

évoqué, s'est appuyé sur ces travaux et sur les propositions de schéma de financement rénové pour faire des propositions ambitieuses et améliorer la qualité du service et l'attractivité pour les salariés du secteur. Ce rapport évoque justement

Nous devrons désormais travailler sur la base du rapport à la meilleure façon de procéder pour que les financements apportés au secteur permettent réellement de mieux rémunérer les personnels et d'améliorer l'attractivité du secteur. Au-delà de ces sujets sur l'aide à domicile, le Gouvernement a indiqué vouloir engager rapidement un grand plan Métiers pour revaloriser tous les métiers du grand âge.

solidarités et de la santé. Monsieur le secrétaire d'État, le 13 septembre 2018, le Président de la République présentait les grandes lignes de la stratégie nationale de lutte contre les « inégalités de destin » et annonçait que 8 milliards d'euros seraient consacrés à sa mise en oeuvre. Je salue plusieurs des initiatives de ce plan, notamment celles qui touchent à la protection de la petite enfance et au soutien apporté aux crèches : ce sont des sujets qui me sont chers et importants pour nos territoires. Toutefois, aucune mention n'a été faite des outre-mer dans ce discours affirmant qu'il fallait « faire plus pour ceux qui ont moins ». La pauvreté y est pourtant bien plus massive qu'en Hexagone puisqu'elle touche une personne sur cinq en Martinique et huit personnes sur dix à Mayotte, Une déclinaison classique du plan est prévue dans les territoires ultramarins comme dans les autres collectivités, mais, au-delà, aucune mesure prenant acte de cette situation particulière ne semble avoir été décidée. Aussi faut-il rappeler que les revenus de solidarité active, dits RSA, versés par les conseils départementaux d'outre-mer ne sont pas compensés par l'État dans leur intégralité. Le nombre de personnes au RSA représente ainsi près de 22 % de la population en Guadeloupe. Si de nouvelles charges sont attribuées aux départements dans le cadre du plan national, il sera nécessaire de prendre en compte les coûts existants. Monsieur le secrétaire d'État, pourriez-vous expliciter les modalités de déclinaison du plan Pauvreté dans les outre-mer ? Des mesures spéciales sont-elles prévues pour ces territoires ?

ou encore de la Guadeloupe, sur la base du volontariat, qui pourra dans les mois à venir faire l'objet d'une convention. Celle-ci traduira l'investissement nouveau de l'État en matière de prévention et de lutte contre la pauvreté, aux côtés du conseil départemental.

avec la prévention des sorties dites « sèches » de l'aide sociale à l'enfance, la création des référents de parcours pour un meilleur accompagnement des RSA, le lancement du premier accueil social inconditionnel et l'amélioration de l'orientation et de l'insertion des allocataires du RSA

La conférence régionale des acteurs se tiendra le 15 avril prochain. Cette rencontre devra permettre une appropriation des enjeux de la stratégie et la mise en place de l'animation de cette stratégie par les acteurs concernés, car c'est bien la spécificité et la force de la méthode

Ensuite, sur la base d'un diagnostic local coconstruit, des priorités seront définies en matière d'enfance, de jeunesse, d'insertion ou d'accès au droit. Nous déploierons les mesures de la stratégie avec l'ouverture de nouvelles places de crèche sur l'île, la création de points conseil budget pour lutter contre le surendettement, le lancement des petits-déjeuners dans les écoles volontaires, la création de centres sociaux, le renforcement des interventions des éducateurs spécialisés, l'aide aux communes pour la tarification sociale dans les cantines, le développement de centres de santé ou encore le déploiement de la garantie jeunes pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Enfin, je vous confirme qu'aucune charge nouvelle ne sera attribuée aux départements. Au contraire, des moyens nouveaux seront apportés aux outre-mer par la stratégie Pauvreté dans l'objectif effectivement de faire plus pour ceux qui ont moins. La parole

par la verrerie de Givors, soit 82 ! C'est énorme. Pourtant, seize ans après la fermeture de cette verrerie, les salariés sont toujours en attente d'un reclassement du site en zone amiantée Ce reclassement permettrait à ces femmes et à ces hommes d'obtenir un certificat d'exposition, de bénéficier d'un suivi post-professionnel et, le cas échéant, de voir reconnaître leurs pathologies comme des maladies professionnelles, accompagnées d'une indemnisation du préjudice d'anxiété pour les expositions diverses.

Monsieur le secrétaire d'État, sur les 645 anciens verriers membres de l'association des victimes, 211 sont décédés et 73 sont aujourd'hui malades. L'âge moyen des décès est de 70,5 ans, soit neuf ans de moins que la moyenne des hommes en France. Douze maladies professionnelles ont été reconnues, mettant en cause l'exposition au benzène, à l'arsenic, à la silice, à l'amiante, aux huiles minérales, aux hydrocarbures et aux solvants.

Dans cette perspective et compte tenu de ces éléments, quand le Gouvernement compte-t-il prendre des dispositions afin de reclasser cette zone mortifère en site amianté ? Ce reclassement, s'il n'a pas le pouvoir de soigner, aurait au moins le mérite d'apaiser la souffrance des victimes et de leurs familles.

de verre creux de la région et de définir les mesures de prévention adaptées, qu'il s'agisse de la formation des personnels à l'usage des équipements de protection individuelle ou d'une meilleure information sur les risques. Ces résultats ont été diffusés auprès de l'ensemble des acteurs de la prévention les entreprises concernées, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puis leur comité social et économique, ainsi que les préventeurs de la Carsat et les équipes des centres de consultations de pathologies professionnelles de la région. Par ailleurs, les anciens salariés du régime général ayant été exposés à des substances ou des procédés cancérogènes pendant leur vie professionnelle peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un suivi médical post-professionnel. Ce suivi, pris en charge par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, est accordé par la Caisse primaire d'assurance maladie sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail. Toutefois, ce qui arrive souvent, dans le cas où l'assuré est dans l'impossibilité de fournir cette attestation, notamment parce que l'entreprise a disparu, l'assurance maladie se chargera de vérifier l'effectivité de l'exposition avant de proposer à l'intéressé le suivi médical adapté. Les anciens salariés des verreries de Givors qui le souhaitent peuvent ainsi prendre contact avec leur caisse afin de mettre en place ce suivi, si tel n'est pas encore le cas. En outre, les salariés et anciens salariés peuvent demander la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie. Ils disposent pour ce faire d'un délai de deux ans à compter du certificat médical les informant du lien possible entre leur maladie et leur activité professionnelle ou à compter de la date de cessation d'activité si elle est postérieure. Enfin, la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 de l'assurance maladie-risques professionnels prévoit d'améliorer l'accompagnement des personnes dans leurs démarches visant à la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie, ayant conscience de l'enjeu. Une expérimentation sera ainsi lancée, d'ici à l'été 2019, pour mieux informer les personnes sur l'origine potentiellement professionnelle de leur pathologie. En outre, l'information sur la procédure de reconnaissance sera améliorée,

d'État, depuis plusieurs semaines, les artisans du bâtiment nous interpellent sur la situation très préoccupante du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale, le Fafcea. Jusqu'en janvier 2018, les cotisations de ce fonds étaient collectées par la direction générale des finances publiques. Ce sont maintenant les Urssaf qui en assurent le recouvrement. Comme vous le savez, cela ne fonctionne pas très bien et le financement de la formation professionnelle des artisans est gravement menacé. Les comptes présentent un déficit de 32 millions d'euros parce que 170 000 adresses d'entreprises ont disparu des fichiers. De 72 millions d'euros en 2017, on passe à 33,8 millions d'euros en 2018, et la collecte a encore diminué d'un tiers en 2019. Je sais qu'une réunion s'est tenue au ministère du travail il y a quelques jours avec les parties prenantes et qu'un rapport de l'Inspection générale des affaires Je sais également que vous avez décidé de reporter le remboursement des avances opérées au fonds d'assurance à 2020 et que des mesures d'urgence sont censées être prises En dépit de ces annonces, les artisans m'alertent sur les engagements financiers du fonds d'assurance, qui sont toujours suspendus, notamment parce que la collecte pour 2019 est très inférieure à vos prévisions. De même, si l'Agefice se dit prête à soutenir la formation des artisans, cela ne se fera pas dans n'importe quelles conditions. Les salariés et les dirigeants salariés sont par exemple automatiquement exclus, si l'on s'en tient aux critères pratiqués par l'Agefice. Monsieur le secrétaire d'État, vous l'aurez compris, la situation manque de clarté et les artisans sont suspendus aux engagements financiers, qui ne sont pas encore clairement définis.

Comme vous le savez, et vous en avez rappelé un certain nombre d'éléments que je vais réitérer devant vous, la collecte de la contribution à la formation professionnelle des artisans est assurée par les Urssaf et non plus par la direction générale des finances publiques, en application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cette modification des modalités techniques de collecte a entraîné des difficultés de trésorerie pour le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale, ainsi que pour les conseils de la formation. Ces difficultés s'expliquent encore par le fait que de nombreux artisans salariés, assujettis à la fois à la contribution à la formation professionnelle en tant que travailleur indépendant versée au Fafcea et à la contribution à la formation professionnelle en tant que salarié versée à leur opérateur de compétences, ont refusé de s'acquitter, à l'automne 2018, de la contribution due en tant que travailleur indépendant, contestant la légalité de ce double assujettissement qui n'existe que pour les artisans. Des mesures ont été prises rapidement par les services de l'État : l'Agence France Trésor a avancé 15 millions d'euros et l'Agence centrale des Des discussions se sont également rapidement engagées avec les chambres de métiers et de l'artisanat pour trouver une solution durable. Ainsi que j'aurai l'occasion de le redire à votre collègue le sénateur Luche, plusieurs réunions ministérielles et interministérielles ont été organisées ces dernières semaines avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment les dirigeants du du Fafcea et les représentants de toute la filière. Ces réunions ont abouti à proposer un certain nombre de mesures d'ordre financier permettant de poursuivre la prise en charge des actions de formation des artisans, et ce sur l'ensemble de l'année. Les versements de l'Acoss au fonds et aux conseils de la formation sont intervenus lundi 18 mars 2019, ce qui permet de traiter la situation sur le court terme. sur le court terme. De plus, un gel des remboursements des avances accordées en 2018 a été décidé et un complément exceptionnel de financement sera apporté en 2019, dont les modalités précises sont en cours de définition. Par ailleurs, vous le savez, une mission de l'Inspection générale des affaires sociales a été lancée pour étudier le système de collecte et de répartition de la contribution à la formation professionnelle entre les fonds d'assurance formation des non-salariés et la situation comptable et financière du Fafcea et des conseils de la formation, afin de trouver une solution pérenne. Le rapport de cette mission sera remis à la fin du mois de juin prochain, afin d'inscrire les propositions qui seront retenues dans la durée, au plus tard le 1 janvier 2020.

plus bénéficier de leur droit à la formation. Pourtant, ces artisans restent prélevés de leurs cotisations. Surtout, dans plusieurs domaines d'activités, ces formations sont obligatoires pour exercer leur activité et travailler. Quelle est la cause de cette perte du droit à la formation ? Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un problème lié à des changements administratifs ! En effet, la charge de la collecte des contributions à la formation professionnelle des artisans est transférée de la direction générale des finances publiques vers les Urssaf.

170 000 entreprises artisanales répertoriées par le Trésor public ont disparu du fichier des Urssaf. La conséquence est que le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale affiche un déficit de 32 millions d'euros

Aux dernières nouvelles, il semblerait qu'un autre fonds, l'Agefice, vienne temporairement financer la formation des artisans. Cette solution ne peut être que provisoire puisque cet organisme exclut les dirigeants salariés et les salariés des entreprises artisanales.

réaffirmer, s'il en était besoin, à quel point le Gouvernement partage avec vous la conviction que l'artisanat est le tissu économique de proximité qui irrigue tous nos territoires, le savoir-faire à la française dans toute son expression. Ces derniers mois, les actions que le Gouvernement mène pour développer la filière d'excellence qu'est l'apprentissage comme les différentes réformes conduites par Muriel Pénicaud concourent à conforter ces professionnels et à renforcer notre tissu

encore tout récemment. Elles ont abouti à proposer un certain nombre de mesures d'ordre financier pour parer à l'urgence. Comme je le disais précédemment, des versements de l'Acoss au Fafcea et aux conseils de la formation sont intervenus le 18 mars dernier, permettant de traiter la situation à court terme. Parallèlement, un gel des remboursements des avances accordées en 2018 a été décidé et un complément exceptionnel de financement sera apporté en 2019, dont les modalités restent à définir, mais qui permettra d'assurer, à défaut d'un système pérenne, la dispense la dispense des formations sur l'année 2019. Je rappelle à la Haute Assemblée qu'une mission de l'Inspection générale des affaires sociales portant sur le système de collecte et de répartition de la contribution à la formation professionnelle entre les fonds d'assurance formation des non-salariés et la situation comptable et financière du Fafcea et des conseils de la formation a été lancée, afin de trouver une solution durable. Son rapport sera remis fin juin, pour une décision au plus tard le 1 janvier 2020.

Monsieur le secrétaire d'État, la presse s'est de nouveau fait l'écho, il y a quelques jours, d'une note selon laquelle l'hypothèse d'un détachement progressif des conseillers techniques sportifs du ministère des sports vers les fédérations demeurait largement à l'étude. Une lettre plafond du 26 juillet 2018 émanant du Premier ministre demande en effet une réduction du schéma d'emplois du ministère des sports de 1 600 équivalents temps plein pour la période 2018-2022. Cette lettre précise que le schéma d'emplois reposera sur une transformation du mode de gestion des conseillers techniques sportifs et sur la réduction de leur nombre. Cette perspective continue de susciter une très forte inquiétude dans le milieu sportif. Dès la nomination de Mme la ministre des sports, au mois de septembre dernier, le président du Comité national olympique et sportif français lui a fait part de son opposition au bouleversement d'un « système sur lequel repose en très grande partie l'organisation fédérale Un rapport établi par l'Inspection générale de la jeunesse et des sports a aussi récemment pointé qu'un « scénario de rupture pourrait notamment se traduire par une désorganisation totale du système de performance sportive français », alors que notre pays doit, cent ans après les huitièmes olympiades, accueillir de nouveau les jeux Olympiques. Les auteurs de la mission d'évaluation soulignent « les réelles contraintes juridiques et financières, ainsi que le caractère déstabilisant pour le sport français » d'une telle ambition. Au mois de mars dernier, réunis en assemblée générale, les inspecteurs généraux du sport ont aussi fait part de leur crainte d'une « dispersion d'effectifs déjà réduits, au risque d'une rupture majeure de la continuité du service public de l'État dans le champ du sport Les caractéristiques démographiques actuelles du réseau des conseillers techniques sportifs doivent également nous appeler à la prudence. En effet, sans remplacement des départs à la retraite dans les dix années à venir, ce dernier perdrait 50 % de ses effectifs durant cette période. Monsieur le secrétaire d'État, alors qu'un comité technique ministériel doit se tenir le 16 avril prochain, pouvez-vous nous faire part des axes actuellement retenus par le Gouvernement dans sa réflexion ? La parole est à M. le

dont le caractère public de l'emploi n'apparaît pas toujours nécessaire, à la vie des fédérations et leur permettre de mieux répondre aux attentes des clubs et des bénévoles ». La ministre des sports a, pour sa part, souhaité dès son arrivée engager un travail de concertation, d'écoute et de dialogue sur ce sujet. ce sujet. Elle l'a rappelé récemment lors de son audition devant les députés de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Il est important de le redire : ces agents exercent des missions clés. La rénovation du modèle que nous sommes en train de mener vise à renforcer l'autonomie des fédérations sportives en leur permettant de tirer pleinement parti de ces personnels, dont la compétence et la qualité du travail sont reconnues comme absolument nécessaires au développement du sport français. du sport français. Entraîneurs, formateurs et développeurs expérimentés, les CTS sont devenus des rouages clés du système fédéral et de la réussite de nos sportifs. Rappelons d'ailleurs que c'est au lendemain de la « déroute » française aux jeux Olympiques de Rome que ces agents de l'État ont été placés au sein des fédérations sportives

À l'heure où nous nous projetons vers une organisation plus responsable, plus autonome et plus transparente du mouvement sportif, cette forme d'ingérence de l'État dans la construction de la performance et de la formation paraît caduque. Il s'agit non pas de supprimer les métiers des CTS, mais de revoir les modalités de gestion de ces professionnels.

Évidemment, il n'est pas question de fragiliser les petites fédérations, qui sont souvent des pourvoyeuses essentielles de médailles, mais il importe de trouver un dispositif équilibré permettant aux fédérations de mettre en oeuvre leur stratégie sportive et de déployer leurs ressources humaines de manière autonome. L'État n'a aucune intention de se désengager du sport ; l'évolution du statut des CTS

de Dunkerque. Ce pourvoi faisait suite à l'annulation, par la cour d'appel de Paris, des mises en examen des personnes impliquées dans ce scandale sanitaire, pour la plupart membres de l'ex-Comité permanent amiante, composé d'industriels, de scientifiques et de hauts fonctionnaires. Vingt-deux ans après le dépôt des plaintes, alors que des dizaines de milliers de victimes sont à déplorer, la décision est sans appel pas de procès pénal, car pas de responsables, et encore moins de coupables ! Les juges estiment qu'aucune responsabilité ne peut « être imputée à quiconque », en « l'absence de faute caractérisée » et compte tenu « du contexte scientifique de l'époque et de la méconnaissance des risques encourus encourus ». Faut-il rappeler pourtant que des travaux scientifiques ont démontré, dès les années soixante-dix, les dangers de l'exposition à l'amiante et qu'un rapport sénatorial de 2005 qualifiait le CPA de « lobby de l'amiante », cet organisme ayant fait « le choix de continuer à utiliser l'amiante et de retarder le plus possible son interdiction » Madame la ministre, ce dossier ne peut pas être refermé. L'amiante tue toujours dix personnes par jour et tuera encore pendant de nombreuses années. Beaucoup de personnes se battent pour obtenir ce procès pénal. Il n'est pas possible de continuer à se « réfugier » derrière la séparation des pouvoirs et de se contenter du sentiment du devoir accompli au moyen des indemnisations, aussi justifiées soient-elles. À À ce propos, j'accueille avec satisfaction une autre décision de la Cour de cassation, qui ouvre à tous les salariés ayant été en contact avec l'amiante la possibilité de faire valoir le préjudice d'anxiété. il faut aller plus loin : l'injustice doit être réparée et les responsables doivent répondre de leurs actes. Cela passe par un procès pénal. Je souhaite donc savoir, madame la ministre, ce que compte faire le Gouvernement pour empêcher toute impunité pénale des responsables dans le drame de l'amiante. La

prenant toute la mesure des souffrances des victimes de l'exposition à l'amiante, la ministre de la justice partage la légitime préoccupation de voir les procédures judiciaires engagées en ce domaine traitées avec toute l'efficacité et la célérité requises. Il est vrai que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté, dans deux arrêts du 11 décembre 2018, les pourvois formés par les associations de défense des victimes de l'amiante dans les dossiers de l'affaire de Jussieu et du chantier naval Normed de Dunkerque. Dans le cadre de l'affaire du campus de Jussieu, qui a débuté le 15 novembre 1996, plusieurs personnes physiques avaient été mises en examen des chefs d'homicides involontaires aggravés et de blessures involontaires aggravées, ainsi que trois personnes morales du chef de mise en danger de la vie d'autrui : l'université Paris VI Pierre-et-Marie-Curie, l'université Paris VII Denis-Diderot et l'Institut de physique du globe de Paris. Par arrêt du 15 septembre 2017 confirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassation en décembre 2018, la chambre de l'instruction de Paris a annulé les mises en examen des personnes physiques. Concernant l'affaire du chantier naval Normed de Dunkerque, qui a fait l'objet d'une ouverture d'information judiciaire en 2006, trois personnes physiques avaient été mises en examen.

Ces arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation confirment l'analyse de la chambre de l'instruction selon laquelle il n'existe pas d'éléments suffisants justifiant la mise en examen des personnes physiques précitées en « l'absence de faute caractérisée de [leur] être reprochée du fait de [leurs] fonctions au ministère du travail et de [leur] participation aux activités du [comité permanent amiante],

Un assistant spécialisé a d'ailleurs été spécifiquement recruté pour améliorer le traitement des dossiers de l'amiante. Je vous affirme que la mobilisation du Gouvernement sur ce sujet est entière et n'a d'autre motivation que d'aboutir à une solution humainement acceptable et juridiquement

L'argent et les indemnisations ne font pas revenir les disparus, pas plus qu'ils ne rendent la justice. Il n'est pas acceptable que les responsables n'aient pas de comptes à rendre. Cela dépasse la question de l'amiante. Cette décision de justice est comme un permis de continuer à empoisonner. Je pense au glyphosate ou autres pesticides, par exemple. Rendre justice aux victimes de l'amiante, c'est aussi

Cela aura des conséquences sur l'attractivité de notre enseignement supérieur à l'étranger. Ma question porte sur l'impact de cette mesure sur les jeunes étrangers qui ont effectué toute leur scolarité dans l'un de nos 500 établissements scolaires installés à l'étranger.

L'objectif de la stratégie Bienvenue en France est d'attirer davantage d'étudiants internationaux dans notre pays, francophones ou anglophones, pour leur permettre de s'insérer dans la francophonie.

Vous m'interrogez sur la possibilité de déroger à ces droits d'inscription ou de les moduler lorsque les jeunes ont fait leurs études dans des lycées français. Cela fait partie des discussions que nous avons avec les présidents d'université, ces derniers ayant la capacité, dans la construction de leur stratégie d'accueil et d'augmentation du nombre d'étudiants internationaux, de travailler avec des établissements partenaires et de passer des conventions avec ces derniers. Plusieurs universités se sont déjà engagées à le faire avec un certain nombre d'écoles françaises, et je serai bien entendu très attentive à ce que tous les jeunes qui veulent venir étudier en France aient les moyens d'y être accueillis. Parmi les élèves inscrits dans les lycées français à l'étranger, nous avons effectivement une proportion importante de jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Ils le font néanmoins aujourd'hui majoritairement au sein de classes préparatoires ou d'écoles qui pratiquent des droits d'inscription bien plus élevés que ce que nous prévoyons pour les universités. Il revient donc aux universités de construire avec ces établissements français à l'étranger leur stratégie d'attractivité. La parole Madame la ministre, j'espère que nous pourrons trouver ensemble un compromis. Cela me paraît à la fois nécessaire et juste.

et de l'innovation. Madame la ministre, en tant que membre du groupe de travail « Attractivité des emplois et des carrières scientifiques », qui a pour mission de faire des propositions à votre ministère en vue de la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés rencontrées par les étudiants en double cursus médecine-sciences. Ce cursus permet l'acquisition d'une formation à la recherche et d'un doctorat de sciences au cours des études médicales. L'objectif est de former des cliniciens à la recherche fondamentale, clinique et translationnelle. Grâce à leur double compétence, ces médecins participent à des activités de recherche et jouent ainsi un rôle déterminant dans le développement des innovations cliniques au service des patients. Or, selon une étude de l'association Médecine Pharmacie Sciences, l'articulation entre les formations médicales et scientifiques reste insuffisante. Parmi les problèmes évoqués par les étudiants figure notamment l'organisation actuelle des deuxième et troisième cycles des études médicales, qui, en l'absence d'aménagements, les oblige à interrompre pendant plusieurs années leurs activités de recherche. Les conséquences en sont un taux important de renoncement à la poursuite du parcours de recherche, voire, pour certains, un départ vers des pays valorisant davantage les doubles parcours.

Enfin, les difficultés se prolongent ensuite dans l'aboutissement d'un projet professionnel médecine-recherche, que les seules carrières hospitalo-universitaires ne suffisent pas à combler. Ces éléments expliquent en partie les effectifs relativement faibles des étudiants engagés

madame la ministre,

générale, l'attractivité des carrières scientifiques est un enjeu majeur pour notre pays. Nous partageons cette conviction, et c'est pourquoi j'ai souhaité que vous participiez à l'un des groupes de travail dédié à cette question dans le cadre de la préparation du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Ce groupe de travail a vocation à aborder la question de l'entrée dans la carrière scientifique, et donc de la découverte de la recherche pendant les études, y compris en médecine.

en ville comme à la campagne, l'accès aux activités et sites culturels, ainsi qu'à la pratique sportive. Cet accès est déterminant dans des territoires de ruptures économiques et de précarités sociales. Des bassins de vie dans l'Aisne, la Thiérache par exemple, illustrent cette situation. Aller à la découverte de l'art, favoriser la créativité, ouvrir sur le monde ou d'autres époques, donner confiance en soi, tout cela passe, pour les collèges et les lycées, par l'organisation de sorties pédagogiques. Mais les projets initiés sont confrontés à la problématique des transports dans le monde rural, où la route- le sujet est d'actualité -garde une place incontournable. À Hirson, à la cité scolaire, le conseil d'administration a décidé en décembre 2016 d'acquérir un minibus d'une capacité de neuf places destiné à des déplacements pour la visite d'expositions, des compétitions sportives départementales, voire nationales, des voyages pédagogiques ou encore des forums de lycéens, dans le cadre du programme scolaire de l'année. Pour ces déplacements autorisés par le chef d'établissement, les professeurs, sur la base du volontariat, conduisaient le véhicule avec la couverture d'une assurance tous risques. Or récemment, Mme la rectrice de l'académie d'Amiens a rappelé l'interdiction faite aux enseignants de convoyer leurs élèves, pour quelque sortie que ce soit. En conséquence, des projets ont dû être mis en suspens ou ont vu leur coût fortement augmenter, pénaliser les élèves malgré les initiatives et prises de responsabilité de leurs enseignants. Monsieur le ministre, est-il possible d'envisager une évolution des textes réglementaires visant à donner plus de souplesse, avec l'accord du chef d'établissement et sur la base du volontariat des enseignants, à l'organisation des déplacements à caractère pédagogique ? Une telle évolution bénéficierait d'abord à des établissements de territoires éloignés des métropoles ou des grands centres urbains. contribuerait à faciliter l'ouverture à la culture et à garantir les mêmes chances en milieu rural qu'en milieu urbain. La parole

Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse encourage les sorties scolaires dans la mesure où elles offrent des expériences diversifiées en lien avec les apprentissages. S'agissant du transport des élèves pendant des activités scolaires obligatoires et certaines activités périscolaires les prolongeant, un seul principe prévaut sur les autres, le recours à un conducteur professionnel. Ce principe est précisé dans la circulaire n° 2011-117 du 3 août 2011 relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée. Ainsi, un personnel enseignant ne peut conduire un véhicule personnel qu'à titre exceptionnel, après y avoir été autorisé par l'autorité académique et quand l'intérêt du service le justifie. Il s'agit donc d'une mesure supplétive qui n'est utilisée qu'en dernier recours, c'est-à-dire en cas d'absence momentanée d'un transporteur professionnel ou de refus de celui-ci. Par exception, sous réserve qu'une police d'assurance spéciale soit souscrite, une autorisation permanente d'utiliser leur véhicule personnel pour transporter les élèves peut être accordée aux enseignants et, dans les mêmes conditions, aux personnes privées détentrices de la carte de membre de l'Union nationale du sport scolaire, étant précisé que l'autorisation accordée peut être étendue aux départements limitrophes. Toutefois, le Gouvernement a bien conscience de vos préoccupations liées aux déplacements en milieu rural, où la question du transport reste cruciale. La mise en place de projets pédagogiques se heurte aux contraintes du monde rural, où le moindre déplacement doit se faire en voiture ou en transport collectif, les principaux lieux culturels ou sportifs étant concentrés dans les zones urbaines.

Je vous remercie

par nos collègues de l'Assemblée nationale et sera examiné dans les prochaines semaines au sein de notre assemblée. Les articles 2 à 4 de ce projet de loi traitent directement de l'extension de l'obligation scolaire, actuellement fixée de 6 à 16 ans, dès l'âge de 3 ans. qui concrètement, on le voit, est indispensable. Cette extension du principe fondamental d'instruction obligatoire est une bonne nouvelle pour les plus jeunes de nos concitoyens, notamment pour les familles les plus fragiles ou les plus éloignées de l'éducation. Pour autant, si cette avancée est louable, il est nécessaire de rappeler qu'actuellement 97 % des enfants âgés de 3 à 6 ans sont déjà scolarisés. Il me semble donc que ce projet de loi est l'occasion de conforter à la fois le rôle de l'école maternelle dans les premiers apprentissages des enfants le rôle des enseignants du premier degré. C'est aussi une façon de renforcer les communes dans leur compétence en termes d'accès à l'éducation, comme le définit le code de l'éducation. En effet, l'école maternelle obligatoire, c'est aussi la reconnaissance par l'État d'une équité de traitement avec l'école élémentaire, notamment en termes de remplacement des enseignants, de carte scolaire, d'ouvertures et de fermetures de classes. L'article 4 du projet de loi prévoit que l'État attribuera des ressources aux communes qui justifieront, au titre de l'année scolaire 2019-2020

à contribuer pour les élèves de 3 à 6 ans déjà scolarisés, qui représentent l'immense majorité de cette classe d'âge ? Pouvez-vous aussi nous éclairer quant à la nature de la prise en charge financière par l'État

votre intention. Vous avez appelé l'attention du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire, et plus précisément sur les moyens mis à la disposition des communes pour compenser les surcoûts occasionnés par cette mesure. L'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans correspond à une extension de compétences des collectivités territoriales. En application de l'article 72-2 de la Constitution, une telle extension doit faire l'objet d'un accompagnement financier de l'État. Les modalités de celui-ci seront précisées par un décret en Conseil d'État. L'article 4 du projet de loi pour une école de la confiance prévoit, vous l'avez dit, que l'État attribuera des ressources aux communes qui enregistreraient durant l'année scolaire 2019-2020, et du fait de cette seule extension de compétences, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire 2018-2019. L'augmentation des dépenses obligatoires de la commune s'appréciera au niveau de l'ensemble des dépenses relatives aux écoles élémentaires et maternelles publiques et des dépenses de fonctionnement des classes maternelles ou élémentaires des établissements privés sous contrat d'association. Une fois déterminé, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, cet accompagnement fera l'objet d'un versement annuel pérenne. Il sera versé, selon les situations locales, soit à la commune, soit à un syndicat intercommunal ou à une intercommunalité ayant la compétence de scolarisation. Par ailleurs, concernant les dépenses d'investissement qui seraient occasionnées par l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, elles pourront être inscrites parmi les dépenses prioritaires que le représentant de l'État dans le département peut subventionner dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local, de la dotation de politique de la ville et de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Enfin, compte tenu des perspectives démographiques pour l'ensemble de la population des élèves du premier degré, qui anticipent une baisse de 64 000 élèves à la rentrée 2019, une diminution significative des dépenses obligatoires du bloc communal est à attendre. La parole

Selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, en 2016, un quart des filles de 15 ans ne savaient pas qu'elles possédaient un clitoris et 83 % d'entre elles ignoraient sa fonction érogène. En revanche, elles étaient 53 % à savoir représenter le sexe masculin. Cette méconnaissance n'est pas surprenante ! En France, le corps de la femme n'est jamais représenté intégralement et correctement-

contre lequel l'école doit lutter : c'est un enjeu d'égalité. Le sexe de la femme n'est ni tabou ni honteux. Il faut que les nouvelles générations apprennent, enfin, comment est fait un sexe féminin- les familles ne sont pas toujours à même de transmettre cette information -, en particulier qu'elles sachent situer et comprendre l'organe qui est la source primaire du plaisir sexuel chez la femme. Cette démarche a également des répercussions symboliques. Penser que le vagin est le symétrique du pénis, alors que c'est le clitoris, c'est se tromper au point de croire que les femmes sont dépourvues d'un organe de plaisir. La reconnaissance du clitoris permet donc de sortir de ce schéma sexuel dans lequel les femmes sont en situation de passivité ou de reproduction. Mettre sur un pied d'égalité les sexualités féminine et masculine, c'est lancer les bases d'une sexualité beaucoup beaucoup plus respectueuse du désir et du consentement de l'autre. Reconnaître le clitoris comme un organe de plaisir à part entière, c'est aussi mesurer la portée des mutilations sexuelles dans la volonté de détruire le désir féminin. L'excision est encore très largement pratiquée dans le monde et concerne également la France : l'Organisation mondiale de la santé estime à 180 000 le nombre de femmes risquant l'excision chaque année au sein de l'Union européenne. Je sais que le ministère de l'éducation nationale et

Cet enseignement doit évidemment être adapté à chaque âge de l'enfant, comme le ministère de l'éducation nationale l'a rappelé dans une circulaire du mois de septembre 2018. C'est dans ce contexte de l'enseignement sur le corps humain et dans le respect du développement progressif de l'enfant que l'enseignement sur le clitoris s'inscrit. Concernant la déclinaison de ces programmes dans les manuels scolaires, au nom des principes de la liberté d'édition et de la liberté pédagogique, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse n'intervient pas directement dans le choix des manuels auquel procèdent les établissements. Par ailleurs, vous appelez l'attention sur la question des mutilations sexuelles féminines. Vous avez raison, ces pratiques méconnaissent les droits fondamentaux de la personne, notamment l'intégrité physique et psychologique. Elles constituent l'une des formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces violences sont enracinées dans les inégalités historiques entre les femmes et les hommes. Elles ont des conséquences non seulement immédiates, mais aussi durables sur la santé des femmes. L'engagement de la France dans la lutte contre ces pratiques a été consolidé par la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la Des mesures de sanctions sont prévues par le code pénal et le système judiciaire prévoit également des outils pour protéger les victimes sur le territoire national. Ce cadre légal a été rappelé tout récemment dans une lettre adressée au mois de mars dernier aux recteurs et inspecteurs de l'éducation nationale, afin de renforcer la vigilance de la communauté éducative. En effet, les actions de prévention sur les pratiques de mutilation sexuelle peuvent se conduire à différents niveaux au sein des établissements. Des documents pédagogiques ont été réalisés pour accompagner la formation des personnels et la mise en oeuvre des actions auprès des élèves.

avant le versement des avances ou des aides PAC. La France a déjà obtenu de la Commission européenne une dérogation pour pouvoir verser des avances après les seuls contrôles administratifs, lesquels comprennent les visites rapides.

PAC -avaient été consenties à tous les agriculteurs et payées par l'État. La différence est là. De même, pour préserver l'efficacité des contrôles, il n'est pas possible de prévenir les agriculteurs contrôlés plusieurs semaines à l'avance. En compensation, les avances PAC sont versées de manière régulière pour intégrer les résultats des contrôles au fil de l'eau.

des contrôles administratifs ont lieu. Pour le reste, je suis au regret de ne pas pouvoir répondre favorablement à votre question. Toutefois, je vous indique que je veille comme le lait sur le feu à ce que tout se passe dans les règles de l'art.

un grand quotidien national titrait en première page le 19 mars dernier : « Aides européennes, un fiasco français ». Vous l'avez compris, je souhaite évoquer la situation du programme de septembre 2016, deux ans après le début de la période de programmation, l'association Leader France nous alertait. Deux tiers des conventions n'avaient pas été signés. La désorganisation des régions était principalement pointée du doigt de leur mouvement de fusion et de réorganisation. En 2018, la même association appelait à un plan de sauvetage face au retard accumulé dans l'engagement et le paiement des projets. Les régions, devenues autorités de gestion sans toutefois en maîtriser ni l'instruction ni le paiement, espéraient alors pouvoir résorber le retard. Alors que près de 700 millions d'euros de fonds européens ont été accordés à la France, seuls 13,5 % des fonds ont été programmés à ce jour et 5 % ont été payés en France. Dans le plus récent classement européen, la France se situe en avant-dernière position devant la Slovaquie en matière de consommation des fonds. Dans mon territoire, en particulier pour le Leader du pays de Gâtine, depuis le 29 février 2016, 80 porteurs de projets ont été accompagnés : 67 ont déposé des dossiers, 12 comités de programmation ont été tenus, 36 dossiers ont été validés, mais seulement 14 demandes de paiement ont pu être envoyées en instruction et, à ce jour, 1 seul dossier a été payé ... Alors que 1 614 745 euros ont été alloués au pays de Gâtine, combien pourra-t-il en consommer ? Symboliquement, c'est l'idée européenne qui pâtit de notre incapacité à nous organiser et à bâtir un système efficient aux dépens d'un système administré et nébuleux. On nous dit qu'une année pourrait être accordée en plus pour récupérer ce retard. Quant à la renégociation des nouveaux dispositifs, la France sera-t-elle en mesure de demander de nouvelles enveloppes significatives ? Monsieur le ministre, vous n'êtes pas responsable du circuit de gestion français du programme Leader, mais que comptez-vous faire avec les régions pour sauver durablement le bateau Leader avant qu'il ne finisse par s'échouer ?

Depuis 2014, cela relève de la responsabilité des conseils régionaux, qui ont sélectionné 340 groupes d'action locale et qui ont en charge la sélection et l'instruction des projets. L'État est lui chargé de la production des outils informatiques nécessaires à l'instruction et au paiement.

Aujourd'hui, le rattrapage du retard accumulé relève de la compétence des conseils régionaux. Cette situation illustre bien la nécessaire simplification des responsabilités pour la future PAC. Les services du ministère, que j'appuie, mettent tout en oeuvre avec les régions pour y arriver. Il serait absolument inacceptable de perdre cet argent. J'ai évidemment commencé à discuter et à négocier à l'échelon européen, afin que, pour le cas où nous n'arriverions pas à rattraper l'ensemble du retard,

propres les projets urgents. Tout cela sera-t-il suffisant ? Il est à craindre que de nombreux projets ne restent dans les cartons et que des porteurs de projets ne se trouvent en difficultés. En effet, les règles se sont tellement complexifiées depuis le dépôt de leur dossier ... Oui ! ... qu'ils risquent de ne pas retrouver l'aide demandée au moment du règlement final.